La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du vendredi 30 octobre 2020 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. M. Christophe Priou a fait connaître à la présidence qu'il se démettait de son mandat de sénateur de la Loire-Atlantique à compter du 31 octobre, à minuit. En application de l'article L.O. 320 du code électoral, il est remplacé par Mme Laurence Garnier, dont le mandat de sénatrice a commencé le 1 novembre, à zéro heure. En notre nom à tous, je souhaite la plus cordiale bienvenue à notre nouvelle collègue. Conformément à l'article 1 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, M. le président du Sénat a pris acte de la cessation, le dimanche 1novembre, à minuit, du mandat sénatorial de MM. Sébastien Lecornu et Jean-Baptiste Lemoyne, membres du Gouvernement, qui avaient été proclamés sénateurs à la suite des opérations électorales du 27 septembre 2020. Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, M. le ministre de l'intérieur a fait connaître que, en application de l'article L.O. 320 du code électoral, Mme Nicole Duranton a remplacé, en qualité de sénatrice de l'Eure, M. Sébastien Lecornu en application de l'article L.O. 319 du code électoral, Mme Marie-Agnès Evrard a remplacé, en qualité de sénatrice de l'Yonne, M. Jean Baptiste Lemoyne. Le mandat de nos collègues a débuté le 2 novembre 2020, à zéro heure.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 M. Guillaume Gontard, président du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires demande que le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à la prévention de la consommation illicite et à la réduction du trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs chimiques, et des délits connexes, inscrit à l'ordre du jour du mercredi 4 novembre à seize heures trente, soit examiné selon la procédure normale et non selon la procédure simplifiée. Acte est donné de cette demande. Dans la discussion générale, nous pourrions attribuer un temps de 45 minutes aux orateurs des groupes. Le délai limite pour les inscriptions de parole serait fixé à demain, onze heures. Il n'y a pas d'opposition ? Il en est ainsi décidé. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi organique relatif à la simplification des expérimentations mises en oeuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution

madame, monsieur les corapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour examiner ce projet de loi organique consacré à l'assouplissement des expérimentations.

Le texte que je présente aujourd'hui devant vous répond concrètement aux deux principaux besoins exprimés par les élus et les citoyens ces dernières années quant à l'action publique. Premièrement, le besoin de proximité : la course au gigantisme, qui a marqué la première partie de la décennie 2010, a sans doute laissé nombre de nos concitoyens bien seuls face aux forces de la globalisation, nourrissant ainsi un terrible sentiment de fragmentation pour la Nation et d'abandon pour eux-mêmes. Deuxièmement, le besoin d'efficacité en effet, nombre de territoires font déjà la preuve de leur capacité à s'adapter et à innover pour accélérer les grandes transitions contemporaines- écologique, économique, sociale et numérique des territoires qui montrent d'ailleurs une nouvelle fois, depuis le début de la crise sanitaire, cette grande capacité d'adaptation. Ces derniers mois, plus particulièrement encore ces dernières semaines, j'ai d'ailleurs pu apprécier notre large convergence de vues sur ces sujets. Ici, au coeur de la chambre des territoires, nos nombreux échanges à propos des textes du Gouvernement ainsi que de vos propres propositions ont en effet permis un enrichissement constant, comme en témoignent les amendements déposés sur ce texte. Chacun ayant fait un pas vers l'autre, je constate que les points de divergence sont aujourd'hui minimes. Face aux dynamiques, multiples et complexes, qui traversent en permanence nos territoires et dépassent toujours les cadres institutionnels, le vieux rêve du jardin « à la française »- une place pour chaque chose et chaque chose à sa place -doit en effet être renouvelé. C'est vrai ! Les territoires doivent avoir les moyens d'être plus dynamiques, plus souples, pour répondre aux défis contemporains. Il est temps de reconnaître la formidable inventivité des territoires et de lui permettre de s'exprimer. À nous désormais, au travers de nos politiques publiques, de mieux prendre en compte la diversité et les singularités de leur permettre d'apporter les réponses les mieux adaptées à leurs besoins et à ceux de leurs habitants. C'est ce que j'appelle- c'est l'une de mes antiennes ! -le « sur-mesure », ou le « cousu-main ». Cette nouvelle étape que nous vous proposons aujourd'hui, c'est bien celle d'une décentralisation de liberté et, peut-être plus encore, une décentralisation de confiance : confiance dans les territoires, confiance dans les élus locaux et confiance dans les citoyens. Cette confiance est, je le crois, absolument nécessaire dans le contexte particulièrement difficile que traverse notre pays. À l'heure où nous devons faire face à une crise sanitaire, à bien des égards dramatiques, nous devons également avoir plus que jamais la République en partage. La cohésion des territoires dont je suis chargée impose de marcher sur une « ligne de crête de trouver le point d'équilibre entre la pente naturelle vers davantage de liberté et l'impératif de cohésion nationale, c'est-à-dire d'unité de la République et d'équité entre les territoires. Ce débat est essentiel, et je crois que nous allons avoir l'occasion de l'aborder plus en détail puisque le groupe CRCE a déposé une motion tendant à opposer Le projet de loi organique que je présente aujourd'hui vise à faciliter les expérimentations pour les collectivités locales, afin qu'elles ouvrent la voie à une différenciation durable. Trop d'éléments bloquants demeuraient jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, seules quatre expérimentations ont été menées depuis 2003 sur la base du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution. Le projet de loi organique, issu en grande partie d'une étude du Conseil d'État que nous avions saisi du sujet, doit permettre d'assouplir les conditions des expérimentations territoriales de les rendre, à la fois, plus simples d'accès, plus rapides à mettre en oeuvre et plus attractives pour les collectivités. Premier objectif : simplifier considérablement la procédure d'entrée dans l'expérimentation. Les collectivités qui répondent aux conditions prévues par la loi prévoyant l'expérimentation pourront désormais décider elles-mêmes d'y participer. Vous le savez, elles ne peuvent actuellement qu'en faire la demande, la décision finale relevant du Gouvernement, qui fixe par décret la liste des collectivités admises à participer. L'entrée dans l'expérimentation sera ainsi considérablement facilitée : les collectivités pourront le faire par simple délibération de leur assemblée délibérante, au fur et à mesure qu'elles le décideront. Cette procédure devrait ainsi réduire le délai moyen d'entrée dans l'expérimentation, actuellement d'un an, Les actes pris dans le cadre des expérimentations ne seront plus publiés qu'à titre d'information au, alors que cette publication conditionne aujourd'hui leur entrée en vigueur. le contrôle de légalité sera allégé. Actuellement, tous les actes pris dans le cadre des expérimentations sont soumis à un contrôle de légalité renforcé et dérogatoire, avec un déféré suspensif. ne restreint ce régime spécial qu'à la décision d'entrée dans l'expérimentation, pour éviter que des collectivités ne répondant pas aux conditions prévues par la loi n'entament sa mise en oeuvre. Deuxième objectif : assurer une évaluation plus pertinente des expérimentations. D'abord, le rapport d'évaluation final de chaque expérimentation, transmis au Parlement, est naturellement maintenu. Il s'agit d'un préalable indispensable aux décisions sur le devenir des mesures prises à titre exceptionnel. Ensuite, la commission des lois a introduit un rapport d'évaluation à mi-parcours de chaque expérimentation. J'y suis très favorable. Il s'agirait, en effet, d'un document fort utile pour les collectivités participantes et pour celles qui hésiteraient à rejoindre l'expérimentation.

Ce rapport est non pas un rapport d'évaluation des expérimentations, mais un simple recensement des demandes d'entrée dans les expérimentations. expérimentations. Il n'a plus lieu d'être, dans la mesure où les collectivités entreront désormais directement dans les expérimentations, sans demander l'autorisation du Gouvernement. Troisième objectif, et c'est un élément décisif de notre texte : sortir de l'alternative binaire entre la généralisation ou l'abandon de l'expérimentation. Le législateur aura désormais quatre options à l'issue de la période d'expérimentation

est nécessaire ; la pérennisation et la généralisation des mesures prises à titre expérimental expérimental ; la pérennisation, sans généralisation, des mesures prises à titre expérimental dans les collectivités territoriales ayant participé à l'expérimentation, ou dans certaines

justifiée. Au regard du bilan du dispositif expérimenté, la loi pourra également modifier les dispositions régissant l'exercice de la compétence ayant fait l'objet de l'expérimentation. Il s'agit de laisser au législateur une marge d'adaptation pour effectuer les ajustements nécessaires. Je veux ici préciser que c'est naturellement dans le respect du principe constitutionnel d'égalité que la pérennisation de mesures prises à titre expérimental dans certaines parties du territoire pourra être effectuée. Simplifier ne suffit pas ; il faut aussi accompagner. Pour nous assurer de l'effectivité des futures expérimentations, nous allons renforcer notre organisation institutionnelle pour mieux accompagner les collectivités dans leur mise en place. En premier lieu, nous allons suivre la recommandation du Conseil d'État de créer des « guichets permanents » afin de favoriser ces initiatives. Concrètement, un tel guichet permettra à l'État de recueillir les propositions des collectivités territoriales en matière d'expérimentation, d'expérimentation, et aux collectivités territoriales de solliciter une ingénierie juridique pour les accompagner dans le montage de leurs dérogations aux normes législatives et réglementaires.

lieu, et c'est une constante de notre action depuis 2017, nous renforçons en parallèle l'aide à l'ingénierie pour libérer partout les initiatives et les projets des collectivités.

qu'il donne de nouveaux moyens concrets aux territoires pour imaginer et mettre en oeuvre les nombreux projets et initiatives qui, sans cela, n'auraient peut-être pas vu le jour. Dès janvier 2021, je présenterai en conseil des ministres le second temps de cette nouvelle étape de la décentralisation, avec le projet de loi dit « 3D », ou « 4D » si vous préférez, dans lequel nous allons consacrer les trois principes de différenciation, décentralisation et déconcentration,

Il est guidé par les mêmes grands principes : simplifier- c'est d'ailleurs l'objectif récemment assigné au quatrième « D » que je viens de citer -, accompagner, en rapprochant les moyens de l'État des territoires, et enfin, évidemment, libérer. La parole

en proposant une réforme au souffle plus ardent pour un nouvel élan des libertés locales. Néanmoins, nous voterons ce projet de loi organique, même timide, madame la ministre, modifié par quelques amendements, car force est de constater- et je suis d'accord avec vous -qu'en la matière l'immobilisme est mortifère. Autour de l'expérimentation se noue inévitablement le débat sur la différenciation et l'égalité des droits et des libertés, à laquelle nous sommes tous très attachés. Mais cette égalité des droits et des libertés implique assurément une différenciation de moyens. N'est-ce pas là la raison du droit spécifique aux outre-mer ou aux communes de montagne ?

L'expérimentation rappelle que les théories doivent être observées et évaluées : c'est le prix de la pertinence et de l'efficience, lesquelles sont encore trop éloignées de notre culture. En 2003, un pas audacieux fut accompli avec l'inscription dans la Constitution du droit pour les collectivités de déroger, à titre expérimental et pour une durée limitée, aux dispositions législatives et réglementaires. Vous l'avez rappelé, madame la ministre, à ce jour, à ce jour, seules quatre expérimentations ont été conduites : le revenu de solidarité active, qui a été généralisé ; la tarification sociale de l'eau, étendue dans la loi Engagement et proximité ; les modalités de répartition des fonds libres de la taxe d'apprentissage et l'accès à l'apprentissage jusqu'à l'âge de 30 ans, deux dispositions qui ont été « effacées » ou reprises dans la loi sur l'apprentissage. Le Conseil d'État déclaré que le cadre excessivement contraignant de l'expérimentation expliquait le faible recours à ce dispositif. Deux reproches sont formulés : une procédure trop lourde et une issue binaire,

Vous proposez d'abord, fort pertinemment, de simplifier la procédure, en substituant au dispositif existant une simple délibération de la collectivité, validée après vérification du contrôle de légalité et publiée pour information au. La seconde La seconde simplification porte sur le régime juridique des actes pris par la collectivité dans le cadre de l'expérimentation. Vous souhaitez le rapprocher du droit commun, ce qui est une excellente chose. En effet, la publication au ne serait

Inventer des solutions au jour après jour, c'est le lot quotidien des élus locaux. Osez, madame la ministre, osons leur faire confiance, faciliter leurs initiatives, qui naissent de leur sens des responsabilités, comme on le mesure bien Le Sénat, convaincu de l'impérieuse nécessité d'une nouvelle audace décentralisatrice dans notre République une et indivisible, propose de vous encourager à adopter une démarche

une priorité si l'on veut donner toute l'agilité nécessaire à la mise en place d'expérimentations sur nos territoires, et offrir la capacité à chacune des collectivités de trouver de trouver les ressources et les ressorts nécessaires pour traiter des problèmes spécifiques qui se posent avec une acuité toute particulière sur certains de nos territoires- je pense notamment aux territoires ruraux, dont je suis élu. Enfin,

Alain Marc. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues,

d'une part, les collectivités de même niveau pourraient avoir des compétences différentes ; d'autre part, les collectivités pourraient déroger aux lois et règlements sans passer par la case de l'expérimentation.

de nous présenter un texte constitutionnel accompagnant un texte organique, lors de l'examen récent des propositions de loi pour le plein exercice des libertés locales. Quant au contenu, il n'est pas non plus compatible avec la Constitution dans son état actuel, ce qui justifie

La Constitution consacre plusieurs types d'égalité. Celle qui prévaut entre les citoyens prend son origine dans l'article VI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon lequel la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège,

que nous reconnaissons est celui de la République et ses subdivisions en collectivités sont liées par l'ensemble des principes constitutionnels que j'ai mentionnés.

ajouterait indéniablement de la complexité à un droit déjà peu lisible. Il créerait, en outre, une insécurité juridique sans commune mesure pour les citoyens et pour les élus locaux. Une telle complexification irait à rebours de tout apaisement de la crise démocratique qui touche la France.

Le schéma territorial en ressort émietté et le décideur introuvable. Le Gouvernement a saisi l'opportunité de « faire de la décentralisation » par les élus et pour les élus,

Attribuer une dérogation ou une compétence spéciale à une collectivité revient, en effet, à reconnaître son exceptionnalité et à renforcer un sentiment d'identité particulière. Le statut spécifique attribué à la Corse, en 1991, par exemple, n'a fait qu'exacerber le régionalisme corse.

». Pourtant, ce n'est pas l'identité d'une collectivité qui la rend plus à même de gérer telle ou telle compétence. Enfin, le droit à la différenciation territoriale représente une rupture singulière,

formées autour de métropoles assez puissantes et indépendantes pour se positionner sur le marché de la mondialisation. Le texte qui nous est présenté peut sembler n'être qu'un petit pas

si j'interviens aujourd'hui devant vous pour m'exprimer contre la motion déposée par Mme Assassi et les membres du groupe CRCE, ce n'est certainement pas pour saluer l'ambition et l'ampleur de la réforme du droit des collectivités territoriales traduites dans le texte que nous présente le Gouvernement.

« d'ajustements essentiellement techniques, qui ne sont pas de nature à consacrer un véritable droit à la différenciation

Ce n'est d'ailleurs pas une mauvaise chose, compte tenu des problématiques soulevées, à l'époque, par certaines des orientations territoriales envisagées dans le projet de révision constitutionnelle. Les ambitions affichées du Gouvernement seraient, de toute manière, impossibles à concrétiser par la loi organique. l'encadrement des expérimentations, tel qu'il figure au quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution, impose sur ces questions des limites à la créativité de l'exécutif. Pourtant, le mot d'ordre de « différenciation » a son importance : à une époque où l'échelon local et la proximité sont plus pertinents que jamais dans l'action publique, ce terme résonne chez nos concitoyens et leurs élus locaux. On devine dans le texte d'aujourd'hui un premier pas dans cette direction, dans l'attente d'une loi 3D- ou 4D, entend-on dire aussi maintenant -dont la genèse a été jusqu'ici assez difficile. En l'occurrence, il est question, en plus d'un certain nombre de mesures purement procédurales et de contrôle parlementaire, de rendre plus flexible l'issue des expérimentations, en autorisant la pérennisation locale des dispositions expérimentales, ou leur extension à une partie seulement des autres collectivités. Je comprends la nature des questions juridiques soulevées par Mme Assassi, qui nous dit qu'une telle disposition constituerait une brèche dans les principes d'égalité entre les collectivités, d'une part, et entre les citoyens, d'autre part. En examinant la question sur le plan juridique, je considère néanmoins que les inquiétudes sur la constitutionnalité des modifications qui nous sont présentées restent globalement infondées.

différences ne portent guère de risques pour l'unité nationale de notre pays. Des territoires aussi variés que la Polynésie, la métropole de Lyon ou encore l'Alsace-Moselle- Moselle que je représente au Sénat -possèdent déjà certaines spécificités, sans que cela semble annoncer la fédéralisation de la France. Par ailleurs, comme je le mentionnais, il semblerait que la transition du véhicule constitutionnel au véhicule organique, pour les mesures proposées par le Gouvernement, se soit également accompagnée d'une diminution sensible de leur ambition. Le Conseil Le Conseil d'État, dans son avis du 16 juillet dernier, n'a pas soulevé de difficultés particulières à je me dois aussi de relever que la commission des lois a effectué un travail de consolidation juridique de nature à garantir la constitutionnalité des dispositions de l'article 6 du texte

Une révision du dispositif des expérimentations de l'article 72 de la Constitution, même d'envergure limitée, est un petit pas dans la bonne direction. Dans ses cinquante propositions pour le plein exercice des libertés locales, la Haute Assemblée a déjà posé des jalons. De nombreux travaux restent à mener pour trouver les bons équilibres,

Pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains est en désaccord avec la motion des membres du groupe CRCE, et votera contre.

qui respecte le principe d'égalité des collectivités territoriales ; qui nous a déjà permis d'adopter des dispositions pour certaines communes, dans

dans son avis du 7 décembre 2017, et dans son étude sur les expérimentations, publiée en octobre 2019 : la différenciation est possible à cadre constitutionnel constant et se fonde sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel, plus précisément la décision du 6 mai 1991, laquelle « le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ». Il en résulte donc que les règles régissant l'exercice des compétences locales peuvent être différentes selon les territoires, sous réserve qu'elles soient justifiées par des différences de situation entre ces territoires. C'est la raison pour laquelle le Conseil d'État a permis que nous prévoyions que les mesures prises à titre expérimental puissent être maintenues dans tout ou partie des collectivités expérimentatrices, et étendues à d'autres. Quant à vos craintes que ce projet de loi organique mette à mal l'égalité entre les territoires et l'unicité de la République, je veux faire preuve de la plus grande clarté. D'abord, il est important de distinguer l'égalité « formelle », à laquelle vous faites référence, de l'égalité « réelle Ces dernières années, l'égalité formelle de traitement entre les territoires n'a pas contribué à résorber les fractures territoriales. Au contraire, ces dernières se traduisent très concrètement par de très fortes assignations à résidence et d'insupportables inégalités de destins, ce qui remet fortement en cause notre modèle social.

Voilà pourquoi l'égalité devant la loi doit parfois être contrebalancée par un principe d'équité. En effet, qui comprendrait qu'on traite exactement de la même manière un quartier politique de la ville ou un quartier d'affaires ? Un territoire urbain ou un territoire rural

Le droit français a progressivement fait une place assez large aux expérimentations. C'est ainsi qu'en 2003, après la révision constitutionnelle, le législateur a permis aux collectivités territoriales de déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités- une durée de cinq ans, renouvelable une fois, pour une durée maximale de trois ans -aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences. Cette forme d'expérimentation locale est inscrite au quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution. Les modalités de ces expérimentations ont été précisées par la loi organique du 1 août 2003 relative à l'expérimentation par les collectivités territoriales, dont les dispositions ont été codifiées dans le code général des collectivités territoriales. Toutefois, on peut déplorer que cette forme d'expérimentation n'ait pas prospéré, puisque seules quatre expérimentations ont été menées sur son fondement : l'expérimentation concernant la répartition des fonds non affectés de la taxe d'apprentissage, qui a été abandonnée à la suite de la réforme de l'apprentissage, et celles qui concernaient le revenu de solidarité active (RSA), la tarification sociale de l'eau et l'accès à l'apprentissage jusqu'à l'âge de 30 ans, généralisées avant même leur évaluation. Le faible nombre d'expérimentations menées sur le fondement de l'article 72 de la Constitution ne doit pas nous inciter à penser que les collectivités territoriales sont réservées à l'idée d'utiliser la méthode expérimentale,

dans la perspective de la révision constitutionnelle, nos collègues députés Jean-René Cazeneuve et Arnaud Viala ont estimé que vingt-huit expérimentations mises en oeuvre sur le fondement de cet article concernaient les collectivités territoriales. Le faible recours aux expérimentations locales s'explique plutôt par un cadre excessivement contraignant. C'est d'ailleurs ce qu'a relevé le Conseil d'État dans une étude sur les expérimentations publiée en octobre dernier, dans laquelle il formule notamment deux reproches. Premièrement, la procédure est trop lourde deuxièmement, les issues de l'expérimentation sont binaires : généralisation à l'ensemble des collectivités ou abandon. Aussi, je me réjouis que la commission des lois ait clarifié les issues possibles au terme de l'expérimentation et en ait renforcé l'évaluation, consubstantielle à la méthode expérimentale. Ainsi, alors que le Gouvernement avait indiqué souhaiter se concentrer sur l'évaluation finale des expérimentations, la commission a consacré, conformément aux recommandations du Conseil d'État, trois moments d'évaluation au cours d'une expérimentation l'évaluation finale, déjà prévue dans le projet de loi organique ; une évaluation intermédiaire afin, le cas échéant, d'adapter la mise en oeuvre de l'expérimentation ; et un rapport annuel, qui listerait, d'une part, les collectivités ayant décidé au cours de l'année écoulée de participer aux expérimentations en cours, et, d'autre part, les demandes d'expérimentations adressées par les collectivités au Gouvernement. Par ailleurs, je rejoins la position de la commission, qui a souhaité, d'une part, préciser que la pérennisation sur une partie seulement du territoire se fera dans le respect du principe d'égalité, conformément au cadre constitutionnel en vigueur, et, d'autre part, maintenir l'abandon parmi les issues possibles de l'expérimentation mentionnées à l'article L.O. 1113-6 du code général des collectivités territoriales. Madame la ministre, chers collègues, ce texte permet de procéder à une simplification, certes timide, du recours aux expérimentations locales et prévoit de nouvelles issues au terme de celles-ci.

Monsieur le président, madame la ministre,

Pour encourager les collectivités à recourir davantage à l'expérimentation, l'assouplissement de la procédure permettant d'y participer ne suffira pas ; nous devons également accroître les moyens des collectivités afin de sécuriser, en amont, la méthodologie utilisée et de permettre une meilleure capitalisation des expériences menées.

Nombre d'expérimentations souffrent encore de carences méthodologiques : objectifs contradictoires, faible association des citoyens et des publics concernés par l'expérimentation ou encore absence d'outils d'évaluation. Certaines actions sont également présentées à tort comme des expérimentations, faute de cadre méthodologique et d'évaluation, et ressemblent plus à des manoeuvres visant à faire accepter une décision déjà prise plutôt qu'à une vérification de la pertinence d'une réforme envisagée.

le renforcement du besoin d'ingénierie et d'accompagnement par l'État, l'amélioration des modalités d'évaluation ou encore la capitalisation des expérimentations menées. Enfin, ne l'oublions pas- le Conseil d'État vient de nous le rappeler -, le « recours accru aux expérimentations [ ...] est aussi un symptôme de la complexité et de la rigidité de notre système normatif. mesure où les lois et règlements sont trop nombreux et trop complexes et qu'ils laissent peu de place au pouvoir réglementaire local, nous pouvons assouplir le processus du recours aux expérimentations, mais nous devons aussi veiller à simplifier le cadre normatif et à accélérer les étapes de la décentralisation, de redonner plus de pouvoir aux collectivités locales. La

les principes fondamentaux de la République et du service public. Le présent projet de loi organique définit un cadre élargi en facilitant le lancement de la procédure d'expérimentation,

de faire une République largement différenciée, dans laquelle les principes du service public dû aux citoyens ne seraient pas les mêmes d'une région à l'autre, d'un département à l'autre. Nous devons garder ce

Le savant s'instruit chaque jour par l'expérience ; par elle il corrige incessamment ses idées [ ...], ses théories, les rectifie pour les mettre en harmonie avec un nombre de faits de plus en plus grands, et pour approcher ainsi de plus en plus de la vérité. » Ces mots doivent entrer en résonance avec le projet de loi organique aujourd'hui en discussion. Les réformes incessantes de la décentralisation, depuis 1982 jusqu'au projet de loi 3D annoncé par le Gouvernement, nous montrent comme la vérité peine à se révéler en cette matière. Elles soulignent comme notre droit et nos institutions peinent à être en harmonie avec les faits, lorsqu'il est question de la vie de nos territoires locaux et de nos concitoyens. Face à un tel constat, la possibilité de procéder à des expérimentations locales telles que permises par la Constitution depuis 2003 aurait dû être une source de solutions pour davantage de pragmatisme et une meilleure adaptation du droit. Ce dispositif devait permettre aux collectivités territoriales de déroger, dans le cadre de leurs compétences, sur une habilitation propre et pour une durée déterminée, aux dispositions législatives ou réglementaires existantes, afin d'éprouver la pertinence des réformes envisagées. dispositif, indéniablement prometteur dans ses principes, connut pourtant un succès plus que limité. Cela a pu être souligné, outre le faible nombre d'expérimentations effectuées, celles qui furent menées le furent le plus souvent sans respecter la méthodologie prévue par le constituant. Légitimement, il faut s'interroger sur les raisons de l'échec du dispositif. Est-ce dû à un manque d'intérêt de la part des collectivités territoriales pour ces expérimentations ? Ce n'est pas mon sentiment.

Le faible entrain pour les expérimentations locales est-il alors dû à la contrainte juridique excessive du dispositif en vigueur ? Cette explication n'est sans doute pas suffisante, mais elle peut être avancée et elle justifie qu'il faille en réformer le régime. En effet, cet échec, quels qu'en soient les motifs, est regrettable et nous impose d'y remédier. Des expériences locales seraient l'occasion d'observer les différences que peuvent introduire les territoires dans leur réglementation. Faut-il administrer une zone « hyper-urbanisée » comme on administrerait un territoire « hyper-rural » ? Notre regretté collègue, Alain Bertrand, avait souligné l'attention singulière dont cette « hyper-ruralité »

Face à cela, les zones hyper-urbanisées, telles que les métropoles, sont confrontées à d'autres problèmes politiques : pénurie de logements, habitats insalubres, congestion de la circulation urbaine, concentration des inégalités, densité démographique Face à cet éventail de particularismes, chaque région, chaque département, chaque commune connaît ses propres dynamiques, ses propres problématiques et quand, d'aventure, leurs problématiques sont les mêmes, il est rare qu'elles trouvent des réponses identiques d'un territoire à l'autre, d'une collectivité à l'autre. Pour ces raisons, mes collègues du groupe du RDSE et moi-même sommes favorables à tout mécanisme qui participerait à ce que l'action publique s'adapte mieux aux besoins spécifiques du lieu où elle est mise en oeuvre. L'assouplissement et la simplification du régime juridique des expérimentations locales nous paraissent s'inscrire Toutefois, si ce texte devait constituer un préambule au futur projet de loi 3D, nous veillerions à rester mesurés dans notre approbation, car il ne faudrait pas non plus que les réformes participent à un délitement de l'administration locale sur le territoire national. L'unité républicaine passe aussi par le maintien d'une forme d'uniformité de l'action publique sur tout le territoire. Le réseau des préfectures et des sous-préfectures ne doit pas être délaissé, afin de pouvoir accompagner les collectivités territoriales et favoriser l'accès aux services publics. La Nation française n'est pas un agrégat de collectivités mises bout à bout. Il faut donc veiller à ce que cette différenciation ne conduise pas à un abandon, par l'État et dans l'État, des collectivités locales les plus démunies, les moins armées tant financièrement qu'humainement, pour faire face aux difficultés qu'elles rencontreraient.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, collègues, je tiens tout d'abord à balayer un faux problème, un faux débat, s'il en était encore besoin. Bien évidemment,

ce texte visait déjà à faire plus que simplifier la demande d'évaluation et le contrôle du Parlement sur ces expérimentations. Cela a déjà été dit, mais je tiens à le répéter, vouloir vouloir trop réduire l'évaluation n'est pas un gage d'efficacité. Si l'on cherche à simplifier, c'est bien pour permettre aux élus locaux d'être plus efficaces dans leur prise de décision ; or, justement, nous pensons à l'inverse

qui permet aux collectivités territoriales de déroger, pendant un temps limité et sur un objet circonscrit, aux dispositions législatives et réglementaires régissant l'exercice de leurs compétences.

dangereuse et qu'elle est pertinente. Ainsi, l'idée d'expérimentation renvoie plutôt à une technique d'élaboration des normes fondée sur l'expérience et sur l'évaluation ; elle se distingue donc de la différenciation.

Républicain n'est pas, par principe, hostile à la démarche expérimentale en tant que telle. D'ailleurs, l'expérimentation existe dans de multiples textes : elle concerne les modes d'organisation de la fonction publique ou le transfert de certaines compétences

ne sont pas forcément identiques pour toutes les collectivités qui relèvent de la même catégorie. Je rappelle juste que l'identité ne saurait forcément conduire à l'égalité et qu'il faut traiter de façon différente les situations qui ne sont sens des deux issues ajoutées par le Gouvernement : le maintien des mesures dans les collectivités locales de l'expérimentation pour certaines de ces collectivités ou pour d'autres ; la modification des dispositions régissant l'exercice de la compétence qui a fait l'objet de l'expérimentation. Pour autant, si, je le répète, le texte n'est pas mauvais, va-t-il apporter des solutions à la faiblesse des expérimentations ? Les rend-il plus incitatives ? Rien n'est moins certain. L'exposé des motifs indique que la loi organique permettra d'« illustrer le principe de différenciation territoriale ». Or le texte n'a absolument pas cette portée ! Outre la différence que j'ai soulignée entre expérimentation et différenciation, sans modification constitutionnelle, le projet de loi organique n'a pas la portée qu'il prétend avoir.

le maintien de la possibilité d'abandon, qui était nécessaire. Je répète qu'elle a également insisté sur le fait que l'évaluation est consubstantielle de l'expérimentation. Je crois qu'il faut se réjouir de cette prise de position, parce que la vision du Gouvernement en la matière était trop limitative. Au final, ce texte ressemble surtout à un texte d'attente pour faire patienter les territoires. Qu'y manque-t-il ? Ce n'est

de loi organique d'un autre véhicule juridique qui vous permette de traiter tous ces aspects ? Vous savez que la question de l'ingénierie est discriminante. Vous savez aussi qu'il faudrait sans doute que dispose explicitement de la mission d'inciter à l'expérimentation. Vous savez aussi qu'il manquera des moyens ... Pourquoi ne pas avoir « accompagné » l'ensemble du texte de mesures qui permettent de le rendre opérationnel ? En conclusion, que déduire ? D'abord, par ce texte, l'exécutif envoie deux messages, peut-être à son insu. Il nous annonce qu'il n'y aura pas de révision constitutionnelle jusqu'à la fin du quinquennat, pour l'expérimentation comme pour le reste.

les impôts de production sont toujours supprimés. Je rappelle encore que le plan de relance procède d'une vision centralisatrice, les élus étant amenés avant tout à accompagner le préfet.

nous le voterons. Il ne mérite ni excès d'honneur ni indignité, mais nous resterons dubitatifs quant aux effets qu'il aura dans le temps.

le présent projet de loi organique, comme son intitulé l'indique, a deux objectifs attendus par de nombreux élus : simplifier et différencier l'application du droit. Comme cela a été rappelé, l'expérimentation a été créée par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, qui visait à donner des moyens normatifs à l'organisation décentralisée de la République. Ainsi, le quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution permet aux collectivités territoriales ou à leurs groupements de déroger, lorsque la loi ou le règlement l'a prévu, « à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences ». Cette possibilité offerte aux collectivités territoriales a montré à de rares reprises son efficacité, comme ce fut le cas pour le revenu de solidarité active, la tarification sociale de l'eau, l'accès à l'apprentissage jusqu'à l'âge de 30 ans ou encore la répartition de la taxe d'apprentissage. Alors que la tradition centralisatrice de l'État pèse toujours sur la mise en oeuvre des politiques publiques, l'expérimentation était considérée, à l'origine, comme une façon de renforcer la décentralisation, en donnant plus d'autonomie aux collectivités locales. Aujourd'hui, elle apparaît comme un moyen, souhaité par de nombreux élus locaux, de différenciation des territoires les uns par rapport aux autres. La volonté du Gouvernement de simplifier le recours à l'expérimentation pour assurer plus d'agilité locale, donc plus de différenciation, est louable. Cependant, l'adoption du projet de loi organique avant le projet de loi plus fondateur- du moins l'espérons-nous -et tant attendu « 3D+ » ou « 4D », qui doit fixer l'objectif de différenciation, relève, selon nous, d'un illogisme législatif. Plus clairement, cela consiste à « mettre la charrue avant les boeufs », comme on le dit en pays cauchois, en définissant les moyens avant de connaître clairement la cible. Cela est d'autant plus vrai que, pour donner véritablement tout son sens à l'expérimentation locale, c'est non seulement la loi loi organique qu'il fallait modifier, mais aussi, comme cela a été dit à plusieurs reprises, notamment par les corapporteurs, la Constitution elle-même, ainsi que l'a proposé le Sénat, afin d'éviter le couperet du principe d'égalité pour la pérennisation des expérimentations. Je veux ici saluer l'excellent travail des corapporteurs, Françoise Gatel et Mathieu Darnaud, qui portent, au cours des débats successifs, les propositions du Sénat, sur l'initiative de son président, Gérard Larcher, « pour une nouvelle génération de la décentralisation » et qui tentent ici, par leurs apports, de donner plus de souffle à cet outil technique qu'est l'expérimentation.

de la Constitution, comme le dispositif « territoires zéro chômeur de longue durée », en cours de discussion. Ce demi-échec s'explique par la lourdeur de la procédure, les débouchés limités et l'absence d'évaluation utile. Le principal facteur limitant l'expérimentation territoriale est identifié : la complexité et la lourdeur de la procédure pour pour participer à une expérimentation sont de nature à dissuader toutes les collectivités territoriales de se lancer dans ce projet expérimental. Les sept étapes étapes préalables à l'expérimentation ont surtout conduit à refermer le droit qui avait été ouvert. La simplification des conditions de participation est donc essentielle pour permettre son effectivité.

Mais la multiplication du recours aux expérimentations ne dépendra pas uniquement de la simplification des procédures. Elle dépendra surtout de la capacité de l'État décentralisé à accompagner les projets. Cela impose un changement de logiciel des services de l'État, qui doivent non pas se limiter à contrôler les actes des collectivités locales, mais bien accompagner les élus locaux dans leurs décisions, puisque, aujourd'hui, c'est encore au niveau national, à Paris, que se trouve la compétence pour autoriser ou non une collectivité à participer à une expérimentation. Cette méthode témoigne d'une philosophie de l'État à l'égard des collectivités territoriales qui ne se fonde pas sur une confiance mutuelle, alors que seule la proximité peut permettre une efficience des politiques publiques. Il faut, sur le modèle du tandem préfet-collectivités qui a été réclamé au début de la crise sanitaire, en mars dernier, une organisation opportune pour fluidifier les conditions de leur mise en oeuvre, d'autant que les plus petites collectivités ne disposent souvent ni de l'ingénierie ni des moyens financiers suffisants pour mener seules ces expérimentations souhaitées. Par ailleurs, si la procédure est un frein majeur, elle n'est pas l'unique problème de ce blocage législatif reste celui de la finalité de ces expérimentations. Les expérimentations aboutissent, à la fin des fins, soit à un abandon pur et simple, partout et pour tous, soit à une généralisation nationale sans distinction réelle et territoriale. L'alternative entre abandon et généralisation est brutale et n'incite pas les collectivités territoriales à risquer une expérimentation sans débouchés alternatifs. En proposant que les mesures expérimentales puissent être maintenues dans tout ou partie des collectivités territoriales ayant participé à l'expérimentation et étendues à d'autres, le projet de loi organique ouvre des voies plus attrayantes. Cette possibilité sera ouverte aux collectivités territoriales justifiant d'une différence de situation qui autoriserait qu'il soit ainsi dérogé au principe d'égalité. C'est la logique de cette loi organique, qui, avec les réformes territoriales, dont le Sénat attend beaucoup, doit être le premier pas d'une politique de différenciation territoriale. La différenciation territoriale n'est pas un risque de division. C'est bien une méthode de gouvernance qui permettra de mieux prendre en compte les réalités locales. Nous en avons fait l'expérience avec la loi du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace, qui en est un bon exemple et qui ouvre une voie. Enfin, une bonne expérimentation est une expérimentation évaluée, dont les effets sont mesurés à l'aune des objectifs recherchés. L'évaluation permet de définir les évolutions voulues pour l'expérimentation, tant à son terme qu'au cours de sa réalisation.

De même, l'information chaque année du Parlement est incontournable pour permettre au législateur de connaître les applications différenciées de la loi sur le territoire. En conclusion, nous voterons ce projet de loi organique, qui, même s'il ne consacre pas un véritable droit à la différenciation, lequel mériterait une révision constitutionnelle plus globale, permettra une meilleure agilité dans la mise en oeuvre des politiques publiques, ce que réclament depuis longtemps le Sénat et les sénateurs.

Monsieur le président, madame la ministre,

le texte que nous étudions aujourd'hui est le bienvenu. En effet, il vise à faciliter l'expérimentation, en prévision du très attendu projet de loi 3D. 3D. Voilà qui est bien. Commençons par expérimenter. Nous pourrons ensuite différencier. Je pense que nous ne pourrons avoir une différenciation qu'après une expérimentation réussie. Je veux souligner deux points particuliers concernant ce projet de loi organique : l'évaluation et les moyens mis à la disposition des collectivités pour les accompagner dans ces expérimentations. Premièrement, pour qu'une expérimentation soit réussie- du moins, jugée comme telle -, il est indispensable de faire une évaluation détaillée. C'est sur ce thème que portent principalement les divergences entre votre texte, madame la ministre, et la version amendée de la commission des lois. Un rapport annuel était déjà prévu depuis 2003 pour lister les expérimentations en cours et indiquer les collectivités ayant souhaité réaliser une expérimentation sans en obtenir l'autorisation.

expérimentations en dix-sept ans, dont deux interrompues avant la fin, cela ne justifie pas un rapport annuel ... Mais, à partir du moment où l'on veut vraiment se lancer dans l'expérimentation, et justement avant de mettre en place la différenciation,

ces expérimentations. Le rapport final, quant à lui, permettra de développer cette culture de l'évaluation qui nous manque tant, d'autant que, pour pérenniser les expérimentations, sans passer par une modification

comme l'indique le Conseil d'État, les raisons pour lesquelles, sur le thème expérimenté, la loi peut, à droit constitutionnel constant, différencier les modalités d'exercice des compétences en fonction de différences objectives entre les collectivités territoriales. Cette évaluation permettra à la collectivité concernée de justifier de ces différences objectives. Un rapport intermédiaire vous est également demandé sur chacune de ces expérimentations.

Cela fait beaucoup de rapports demandés par le Sénat qui, d'habitude, n'en est pas très friand, mais j'ai bien entendu, madame la ministre, que vous étiez favorable aux deux rapports d'évaluation- le rapport final et le rapport intermédiaire.

Lors des différentes auditions, je me suis rendu compte que, pour ces différenciations, on évoquait plutôt les départements ou les régions et assez peu les communautés de communes ou les communes. Il est vrai que les expérimentations déjà menées concernaient ces échelles. Il est vrai aussi que l'on ne sait pas de quels types d'expérimentations les collectivités souhaiteront se saisir, mais il est sûr que celles qui réfléchissent à cette possibilité

Sans aller jusqu'aux communes, dont je ne suis pas certaine qu'elles puissent être véritablement concernées par le projet de loi organique, les communautés de communes ou les départements ruraux, souvent plus pauvres et moins calibrés en ingénierie, auront-ils la possibilité de se saisir de cette opportunité opportunité d'expérimenter ? Vous le savez, madame la ministre, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on n'a pas d'idées ... Mais vous m'avez rassurée Mais vous m'avez rassurée : j'ai bien entendu que le guichet unique qui recueillera les demandes aura la possibilité d'accompagner les collectivités sur le plan juridique

sont favorables à ce projet de loi organique, mais ils suivront les recommandations pertinentes de nos corapporteurs de la commission des lois, Mathieu Darnaud et Françoise Gatel. Gatel. Vous savez que nous suivons toujours les recommandations de la nouvelle présidente de notre délégation aux collectivités territoriales ... Les sénateurs du groupe Union Centriste voteront donc la version amendée par le Sénat.

Guy Benarroche. L'amendement tend à inscrire dans la délibération prise par l'assemblée pour s'engager dans une expérimentation le cadre méthodologique qui sera mis en oeuvre. Suivant l'avis des corapporteurs, la commission des lois a adopté le projet de loi organique en précisant les issues possibles à la fin de l'expérimentation et en renforçant son évaluation. Ces deux points participent nettement à l'amélioration du texte initial. Toutefois, un aspect nous semble toujours manquer dans cette nouvelle version : le renforcement du cadre méthodologique

Il s'agit d'ailleurs d'une recommandation du Conseil d'État, qui, dans son rapport, précise que la fiabilité d'une expérimentation dépend largement de la méthode suivie, des conditions de sa mise en place et de son accompagnement. Les conditions de lancement de l'expérimentation ayant toujours un impact sur les résultats produits, il nous paraît indispensable d'inciter le maître d'ouvrage à s'interroger sur les objectifs recherchés et les moyens à atteindre. Renforcer le cadre méthodologique d'une expérimentation est nécessaire à double titre : d'une part, afin d'éclairer les débats au sein de l'assemblée délibérante ; d'autre part, en vue de justifier la dérogation au principe d'égalité, en étant extrêmement précis sur les objectifs recherchés et les moyens mis en oeuvre pour mesurer les résultats produits. La référence au cadre méthodologique dans la délibération de lancement d'un projet existe déjà dans d'autres procédures, par exemple s'agissant des modalités d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal Cet amendement a donc pour objet d'inscrire dans la délibération prise par l'assemblée le cadre méthodologique, à savoir les objectifs, les modalités de pilotage et d'évaluation ainsi que les critères de réussite. Son adoption permettra de garantir les conditions d'une expérimentation réussie.

Néanmoins, il faut veiller à ce que ces expérimentations se déroulent dans des conditions satisfaisantes, afin qu'elles puissent atteindre leur but, celui d'une différenciation territoriale ajustée aux besoins de chaque territoire et de chaque collectivité. Aussi, l'une des principales difficultés qui pourraient résulter du système mis en place par ce projet de loi organique est que la liberté qu'il offre aux collectivités devienne un vecteur d'inégalités. Comment s'assurer que les collectivités les plus isolées, les moins dotées en moyens humains et financiers s'engagent dans les expérimentations avec la même facilité que d'autres plus aisées ? Comment s'assurer que ces collectivités, déjà submergées par les textes, les réglementations et les normes, ne passent pas à côté de cette opportunité d'expérimenter ? La différenciation ne doit pas se faire à plusieurs vitesses. Elle ne doit pas être le privilège de certains territoires. Le législateur doit y veiller à chaque expérimentation, par la mise en place de dispositifs d'aides financières ou de moyens humains ou, plus modestement, de moyens d'information et d'orientation au bénéfice des territoires candidats aux expérimentations. L'objet de cet amendement est donc de poser comme principe que toute loi instituant une nouvelle expérimentation ne se limite pas à dresser une liste des collectivités pouvant y participer : elle devra aussi s'assurer que chaque collectivité puisse effectivement être en capacité de s'engager dans le dispositif expérimental. Quel

est déjà satisfait par les dispositions de l'article L.O. 1113-1 dans leur rédaction résultant de l'article 1 du projet de loi organique. En effet, ces dispositions prévoient que la loi autorisant autorisant une expérimentation précise les catégories et les caractéristiques des collectivités territoriales autorisées à y participer. Bien évidemment,

souligné au cours de la discussion générale, la phase préparatoire au lancement d'une expérimentation est déterminante pour la qualité des résultats produits, donc

Cet amendement vise à supprimer le rapport annuel que le Gouvernement doit transmettre au Parlement, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L.O.

désireuses d'entrer dans l'expérimentation de profiter d'un premier retour d'expérience. Toutefois, et sans surprise, le Gouvernement souhaite, par cet amendement, supprimer le rapport qu'il devrait transmettre au Parlement chaque année et qui m'apparaît aujourd'hui superfétatoire. En effet, l'évaluation à laquelle nous sommes tous attachés est bien garantie à différentes étapes de l'expérimentation. Ce rapport, auquel la commission des lois a dessiné de nouveaux contours, doit désormais présenter les collectivités territoriales participant aux expérimentations. Or il ne semble pas utile que cette information fasse l'objet d'un rapport spécifique, dès lors qu'elle doit déjà figurer dans le rapport d'évaluation établi pour chaque expérimentation. De plus, l'article 2 du projet de loi organique supprime la procédure de candidature des collectivités aux expérimentations, ce qui rend caduc le deuxième objet de ce rapport. Dans un

le Parlement, singulièrement le Sénat, doit s'inviter dans ce débat sur l'expérimentation. Consacrer un rapport annuel sur ce sujet ô combien important,

surprendra donc pas. Nous regrettons qu'un dispositif aussi innovant et aussi important pour l'administration des collectivités territoriales ait laissé de côté l'ANCT. Nous ne doutons pourtant pas que cette dernière puisse jouer un rôle privilégié dans l'accompagnement des collectivités, au titre des différentes expérimentations qui pourraient être développées. ce projet de loi organique est de contribuer à la différenciation territoriale, il faut veiller à ce que cette différenciation soit menée avec le souci constant de l'accompagnement et de l'information des élus locaux comme des administrés.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin est clos.